des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels, supprimé à la suite de la mise en place de la taxe incitative

amendements proposent d'augmenter, au titre de la première année d'application de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le produit de cette taxe dans la limite de 10 % par rapport à l'année précédente. Or un plafond égal au produit de la taxe de l'année précédente a été institué pour la première année d'application, afin de s'assurer que la mise en place de la part incitative ne soit pas l'occasion, d'une manière ou d'une autre, d'augmenter la taxe. En effet, l'instauration de la part incitative a pour seule finalité d'encourager la réduction et le tri des déchets et de responsabiliser les ménages. En outre, le plafond ne s'appliquera pas les années suivantes. Il n'y a donc pas de gel des taux. Par ailleurs, une évolution pouvant aller jusqu'à 10 % du produit de l'année précédente nous semble manifestement disproportionnée

à M. Jacquin ? J'entends la demande d'un lieu de débat spécifique sur le financement de la collecte, de l'enlèvement et du tri des ordures ménagères. C'est un engagement que le Gouvernement peut évidemment prendre,

Mme Christine Lavarde. L'article 20 vise à sécuriser l'assiette de la taxe dite TST-E, due par les éditeurs de télévision au Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel d'octobre 2017 qui en a censuré certaines modalités. Selon l'exposé des motifs du présent projet de loi de finances rectificative, l'objectif de ces modifications est « d'assurer la neutralité de la réforme ». Or il s'avère que les dispositions proposées augmenteraient en réalité le rendement de la taxe. C'est le cas pour les chaînes en diffusion standard, qui voient non seulement leur abattement supprimé, mais aussi leur taux rehaussé de 5,5 à 5,65 %. C'est également le cas pour les chaînes en haute définition, pour lesquelles la baisse du taux

y a quelques jours. La mise en place d'un taux unique de 5,65 % pour la taxe sur les éditeurs de télévision induit des reversements entre acteurs. Les chaînes privées, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5,472 %, verront leur contribution augmenter légèrement, alors que les chaînes publiques, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5,7 %, la verront diminuer

Il faut bien comprendre que la taxe sur les services de télévision est assise non seulement sur les recettes de publicité, mais également sur d'autres recettes, comme la contribution à l'audiovisuel public, les revenus tirés des SMS ou des appels surtaxés, qui, elles, ne font pas l'objet d'un abattement de 4 % et sont soumises au même taux. En réalité, la neutralité de la réforme doit s'apprécier sur l'ensemble de l'assiette de la taxe, afin d'assurer la stabilité des ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ainsi, le taux de 5,65 % a justement été retenu, parce qu'il permet de maintenir le niveau global des ressources consacrées à la politique de soutien au cinéma et à l'audiovisuel

les villes petites et moyennes de province et un certain nombre de centres-bourgs sont aujourd'hui confrontés à de grandes difficultés, en particulier en matière de dynamisation commerciale et de

répondaient à une problématique datée, aujourd'hui en partie dépassée, parce que l'attractivité de ces bâtiments, quelles qu'en soient les qualités patrimoniales, est assez faible d'un point de vue

que la revitalisation des centres-villes passe à la fois par la requalification des espaces publics, la valorisation du patrimoine et la remise sur le marché locatif de logements dans des conditions qui non seulement permettent aux propriétaires et aux investisseurs d'atteindre un équilibre économique,

L'engagement que je prends aura d'autant plus de chances d'être tenu que les appels à manifestation d'intérêt seront organisés au cours du premier semestre de l'année 2018, ce qui signifie

de renforcer la dissuasion d'exploitation des énergies fossiles en alourdissant le barème de la taxe et d'accroître temporairement, tant qu'elles existeront, les ressources financières des départements

Le barème initialement établi prend en compte les caractéristiques géologiques du sous-sol français et son potentiel en hydrocarbures. Il a été calé sur celui des pays voisins, en particulier l'Italie, et est fixé de manière à ne pas remettre en cause l'équilibre économique global.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement a souhaité revoir l'ensemble de la fiscalité minière relative aux hydrocarbures à l'occasion du dépôt du projet de loi mettant fin à la recherche et l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, actuellement en cours d'examen au Parlement. d'hydrocarbures est calculée sur le volume de production annuelle d'hydrocarbures liquides ou gazeux selon des taux progressifs définis par tranches de production. À ce volume de production est affecté un prix de valorisation, prix de vente au départ du champ pour le pétrole et tête de puits pour le gaz, ce qui permet de calculer une redevance en euros. Ces taux sont différents selon la date de mise en service du puits. Si celle-ci est postérieure au 1janvier 1980, les taux sont réduits. Cette redevance n'a pas été modifiée depuis 1981 et maintient une distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et ceux qui Elle ne concernait jusqu'ici que la production d'hydrocarbures et n'avait pas été revue depuis plus de vingt-cinq ans. Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux gisements en mer. Par conséquent, la simplification des taux qu'opère l'article 21 permet d'adapter la fiscalité des hydrocarbures aux réalités économique, énergétique et climatique actuelles. Pour information, en 2013, pour le pétrole,

de cette redevance s'est élevé à 5,5 millions d'euros. L'importante baisse enregistrée par rapport à 2013 est liée à l'évolution du prix du pétrole entre 2013 et 2016. Pour la production de gaz, le barème est constitué de deux tranches. Toutefois, la production de gaz étant quasiment nulle en France depuis l'arrêt du site de Lacq, elle n'a pas entraîné de paiement de la redevance à taux progressif en 2016.

Je vais de nouveau parler de fiscalité et d'écologie. Cet amendement a trait aux réseaux urbains de chauffage et de climatisation très présents à Paris et dans les villes de la petite couronne. Ces réseaux fonctionnent selon deux techniques. première technique fait appel à des tours aéroréfrigérantes situées sur les toits des immeubles : ces tours consomment l'eau de ville pour refroidir les installations et dégagent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. La seconde est la technique dite du qui dérive une fraction d'un cours d'eau sur une faible distance et, dans un délai court, la restitue dans une proportion qui dépasse 99 %. Les installations de sont assujetties à une taxe hydraulique perçue au profit de

de manière à exonérer de nouveau la technique du de la taxe perçue au profit de VNF. Les conséquences sur le budget de l'établissement seraient minimes.

du Gouvernement ? Effectivement, le maintien de l'assujettissement des installations de production d'énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en

La taxe hydraulique est non pas une taxe à visée environnementale, mais une redevance domaniale qui ne peut donner lieu à des abattements au motif que l'usager démontre un comportement plus ou moins vertueux du point de vue de la protection de l'environnement. Cela est en revanche le cas des redevances pour prélèvement d'eau perçues par les agences de l'eau.

Évidemment, les porteurs de projet peuvent le cas échéant en demander la restitution, mais cela signifie alors qu'en cas de recours contre une autorisation connexe nécessaire à la réalisation du projet,

en règle générale, de personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources, équipées d'un appareil de chauffage à charbon et pour qui l'investissement dans un nouvel équipement est hors de portée. Le charbon reste pour eux une énergie bon marché qui leur permet de se chauffer à un coût raisonnable. L'extinction progressive du marché du charbon à usage de chauffage domestique est structurelle et simplement liée à la démographie de ses usagers. Compte tenu du profil de ces consommateurs, la TICC n'a donc aucun effet comportemental et sa forte hausse programmée n'aura qu'un impact punitif qui soulève de forts enjeux de solidarité. le chèque énergie ne couvre déjà pas le montant moyen de TICC pour la consommation domestique annuelle d'un ménage. Cette situation est d'autant plus injuste que le projet de loi de finances pour 2018 a maintenu l'exemption de taxe intérieure de consommation pour les consommateurs particuliers de butane et de propane.

? Cet amendement a déjà été présenté en première partie du

que, lorsque les plateformes en ligne ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, elles appliquent par défaut le tarif correspondant aux hébergements en attente de classement ou sans classement. Il arrive

quant à lui, tend à interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements de verser

vous avez vu, mesdames, messieurs les sénateurs, que le principal opérateur a annoncé, après avoir été reçu au ministère de l'économie et des finances, qu'il retirait son moyen de paiement en France, à la demande du Gouvernement.

en outre, est relativement faible. Airbnb, pour citer ce principal opérateur, a annoncé retirer son système de paiement par cartes prépayées

pendant une période de huit années, correspondant à la durée de l'exonération dont ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui les réseaux câblés, pour ne pas entraver l'accélération des déploiements de fibre optique et préserver une bonne commercialisation, y compris en zone d'initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d'au moins sept ans avec celui de la zone d'investissement privé. Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux de cuivre à celle des réseaux de fibre optique, il est prévu de maintenir cette exonération pour ces réseaux jusqu'à ce que la zone où se situe la prise de la boucle locale cuivre soumise à l'IFER soit labellisée « zone fibrée » au sens de l'article L33-11 du code des postes et des communications électroniques. À cette date, la taxation du FTTH se substituerait à celle du cuivre. Avec un tel système, l'accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France Très haut débit ne seront pas pénalisées.

avec le déploiement du plan France Très haut débit.

Si le statut de « zone fibrée » est effectivement attribué à des zones où l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont déjà avancés, les opérateurs doivent néanmoins encore produire un effort important pour parachever la couverture de ces zones en très haut débit d'ici à 2022 et améliorer la qualité de leurs services.

et ce risque diminue à mesure que les perspectives de rendement deviennent plus certaines. Une prolongation pour trois années supplémentaires paraît donc, à la fois, superflue et coûteuse pour les régions. Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Chaize, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l'avis du Gouvernement

La nouvelle taxe sur la fibre optique aura pour conséquence de restreindre l'accès au numérique dans les collectivités d'outre-mer, dont les besoins en connectivité sont à la mesure de la distance qui les sépare de la métropole.

Le présent amendement tend donc à reconnaître la spécificité des collectivités d'outre-mer, notamment en termes de coûts de construction et d'exploitation de réseaux, en les maintenant hors du champ d'application de cette nouvelle taxe, et à permettre ainsi le déploiement complet du plan France très haut débit dans ces territoires éloignés de la métropole.

Même avis, pour exactement les mêmes raisons.

: La parole est à M. Charles Guené. Cet amendement tend à autoriser le bloc communal à distinguer les dépenses d'investissement de celles de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées. transférées. Il faut permettre cette distinction, car, lorsqu'un transfert de compétences comporte un volume important de dépenses d'investissement, cela peut conduire à un déséquilibre des budgets communaux et il importe que nous ne contribuions pas à dégrader mécaniquement les ratios financiers des collectivités dans ce cadre, surtout dans la

Gouvernement ? Je confirme que cet amendement est satisfait. En application des dispositions de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016, les communes et les EPCI peuvent imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement. Cette imputation peut être décidée dans le cadre de la révision libre du montant de l'attribution de compensation prévue au 1 du V de l'article 1609 C du code général des impôts, c'est-à-dire après délibérations concordantes à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres.

La DSC, qui, à l'origine, était uniquement un outil de péréquation, est progressivement devenue un vecteur de redistribution de ressources à l'intérieur de l'intercommunalité, et il est important qu'on puisse aussi disposer de cette faculté.

dédiée à l'investissement au sein de la dotation de solidarité communautaire revient à créer une sorte de subvention d'investissement dont la répartition ne se ferait pas

générée par cette IFER. Le présent amendement vise à intégrer l'IFER issue des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l'article 78 de la loi de

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est bien conscient des problématiques financières qui concernent les territoires ayant subi ces dernières années la fermeture d'une centrale thermique. L'amendement proposé porte cependant atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales et les groupements

le dispositif actuel de compensation financière prévu par la loi de finances pour 2010 est en principe suffisant pour permettre aux collectivités concernées de bénéficier d'une compensation dans le délai de deux ans suivant la perte effective de ressources fiscales. Cela ne répond pas, monsieur Guené, à votre inquiétude au-delà

il faudrait évaluer ces pertes non seulement en pourcentage des frais de fonctionnement, mais également en valeur absolue rapportée à l'autofinancement de chacune des collectivités. Ce double cliquet serait intéressant. La parole est à M.

THLV, afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et de lutter contre la désertification. Les communes en zone tendue n'ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en oeuvre une THLV. Les logements vacants sont

: la taxe sur les logements vacants étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leurs logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de la

en zone tendue où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l'occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance. Cet amendement ne remet en cause ni la taxe sur les logements vacants perçue par l'ANAH ni le système de plafonnement actuel

l'amendement n° 54 rectifié . Afin de simplifier le régime des communes nouvelles et de ne pas pénaliser leurs contribuables, le présent amendement vise à maintenir les abattements utilisés pour le calcul de la taxe d'habitation issus du transfert de la part départementale au bloc communal en cas de création de commune nouvelle.

car l'harmonisation des abattements peut conduire à une augmentation du montant des cotisations de taxe d'habitation payées par les contribuables. Néanmoins, s'agissant des suites du transfert

qui a été retenue lors de l'examen de la dernière loi de finances rectificative, afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d'homogénéiser leurs politiques d'abattement de taxe d'habitation et ainsi de minimiser l'impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.

: La parole est à M. Patrick Chaize. L'incitation à la création de communes nouvelles a été confortée par le projet de loi de finances pour 2018, avec l'augmentation du seuil de population pour bénéficier des incitations financières, la prorogation de la durée du bénéfice, la bonification de la DGF en cas d'extension de la commune nouvelle, la prolongation de la durée du bénéfice de la DGF bonifiée. Le Sénat a également adopté des amendements tendant à maintenir la dotation de solidarité rurale, ou DSR, en cas de transformation en communes nouvelles, et à conserver le bénéfice par les communes nouvelles de la somme des DSR des anciennes communes qui les composent. Cet amendement s'intègre donc parfaitement dans la démarche d'encouragement et de soutien aux communes nouvelles. Il s'agit de garantir le montant de la dotation perçue au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale. Concrètement, afin d'éviter un effet trop brutal pour les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale, ces dernières percevront au moins 75 % de la somme que chaque commune percevait l'année précédant la fusion des communes. L'antériorité des communes anciennes devient celle de la commune nouvelle. Rappelons enfin que les communes nouvelles sont constituées des actifs et des passifs des anciennes communes. Quel est l'avis de la commission ?

de l'ensemble des communes membres d'un EPCI et qui ont ensuite adhéré à un autre EPCI ont été pénalisées, car les produits intercommunaux des EPCI absorbés n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'effort fiscal agrégé de leur ensemble intercommunal. le présent amendement tend à corriger cette anomalie en prenant en compte dans le numérateur de l'effort fiscal agrégé les produits anciennement perçus par le ou les EPCI absorbés à la suite de la création d'une commune nouvelle.

collègues, il existe trois modalités de répartition du FPIC au sein d'un ensemble intercommunal : la fameuse répartition de droit commun, qui prend en compte le potentiel financier par habitant et la population ; une répartition libre qui est décidée à l'unanimité

une répartition dérogatoire, qui peut être décidée à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI. Dans ce cas, il a été prévu que cette répartition dérogatoire ne peut pas conduire à s'écarter de 30 % de la répartition de droit commun. Vu les règles de majorité- deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI -, ce garde-fou est nécessaire pour s'assurer qu'une ou plusieurs communes ne se retrouvent pas, contre leur gré, à devoir par exemple supporter un prélèvement trop important.

des procédures engagées par des collectivités et des établissements publics dans le cadre du fonds de soutien créé par la loi du 29 décembre 2013 pour répondre à la catastrophe connue liée aux emprunts structurés. structurés. Ils répondent au cas très spécifique de collectivités qui avaient demandé l'aide du fonds de soutien dans les délais prévus pour plusieurs dossiers distincts et qui ont conclu une transaction dans le cadre du fonds de soutien

a parfois manqué lorsque plusieurs dossiers étaient concernés, au regard de la complexité des négociations engagées avec plusieurs établissements distincts de manière simultanée et dans un cadre très souvent confidentiel du fait des contentieux encore en cours avant les transactions. Il s'agit là non pas d'une réouverture du fonds de soutien ni de nouvelles demandes, mais d'une prolongation du délai d'obtention très circonscrite pour des collectivités qui avaient déjà déposé un dossier dans le délai prévu par la loi, à savoir le 30 avril 2015. Cette mesure ne créerait aucune injustice par rapport à des dossiers qui n'auraient pas été déposés dans les délais ni aucun risque juridique pour le dispositif global du fonds de soutien elle n'aurait aucune incidence sur les dépenses de l'État. Nous proposons simplement de parfaire le dispositif initialement instauré pour permettre au maximum de collectivités qui avaient démontré leur volonté de sortir de ces emprunts d'en bénéficier.

était assez clair : à compter de la notification de la décision d'attribution, l'ordonnateur dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l'État dans le département. Pourquoi certaines collectivités

du Gouvernement ? L'examen de ces amendements me permet de rappeler que le fonds a permis de résoudre les difficultés de près de 580 collectivités, pour un montant de 2,56 milliards d'euros, ce qui démontre aussi son efficacité. vous proposez la réouverture du fonds de soutien destiné aux collectivités ayant déjà déposé un dossier avant le 30 avril 2015 et qui ont accepté l'aide de ce fonds au titre de certains emprunts et l'ont refusé pour d'autres. Cette date limite avait été fixée après une longue concertation avec les collectivités concernées, et aucune demande intervenue après cette date n'a été instruite et ne peut être prise en charge, afin de respecter un principe d'égalité de traitement entre les collectivités. La réouverture ou la prolongation, selon la façon dont on envisage les choses, ne peut pas être retenue par le Gouvernement.

Ce rapport permettra d'analyser les modalités d'évaluation des établissements industriels, les différents cadres de qualification et leur impact. De plus, vous en conviendrez, cette question pourrait être abordée dans le contexte plus large des assises de la fiscalité agricole. En outre, je vous rappelle que, dans l'attente de la remise du rapport précédemment évoqué, le

En cohérence avec les dispositions de l'article 24, le présent amendement tend à réduire le taux de la taxe sur les bonis dus par les entreprises d'assurance de dommages dans les mêmes conditions que celui de l'intérêt de retard, auquel il se rattache. De tels ajustements ont déjà été opérés par le passé.

des dossiers des non-résidents. Seulement, voilà, depuis juillet dernier, la DRESG est devenue la direction des impôts des non-résidents, la DINR. Elle s'est vu retirer certaines tâches de nature administrative que cet article entend opportunément confier aux deux autorités indépendantes précitées.

que la grande vague de réduction de l'emploi public ne frappe à son tour la DRESG, devenue DINR, et que quelques postes ne disparaissent encore à cette occasion

actuelle, un groupement d'intérêt public, ou GIP, assume pour le compte de l'État la gestion des systèmes d'enregistrement des demandes de logements sociaux. Ce GIP est présidé par l'Union sociale pour l'habitat.

et qu'elle doit être principalement consacrée à la réalisation d'activités industrielles. Le critère d'autonomie est celui qui est prévu à l'article 11 de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l'entreprise. enfin, compte tenu des modifications qu'appelle pour les entreprises la mise en oeuvre de ces nouvelles règles- je songe par exemple à la révision des contrats de fourniture d'électricité -, un délai d'entrée en vigueur de six mois est ménagé.

présenter l'amendement n° 138 rectifié . L'exonération de contribution au service public de l'électricité, ou CSPE, prévue par l'article 266 C du code des douanes transpose la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l'électricité, d'exonérer de taxe l'électricité produite par les petits producteurs. Cet amendement tend à compléter l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale visant à revenir à la pratique des douanes : appliquer l'exonération uniquement en cas de consommation intégrale.

selon un calendrier s'échelonnant entre juin et novembre 2017. Dans ce cadre, cet amendement tend à autoriser les collectivités territoriales à accéder directement au système d'immatriculation Cette mesure revêt de nombreux avantages. Elle permettrait d'abord de délivrer automatiquement une carte de stationnement résidentielle dès l'enregistrement du véhicule. Les automobilistes n'auraient plus besoin d'apporter une copie de leur carte grise ; il s'agit donc d'une simplification administrative pour les usagers. L'accès au SIV pourrait également servir à mettre en place de nouveaux tarifs de stationnement en fonction des préoccupations préoccupations des collectivités. Celles-ci pourraient ainsi inciter les usagers à utiliser des véhicules moins polluants en choisissant des critères spécifiques pour ces tarifs, comme le type de motorisation ou le nombre de chevaux fiscaux. Toujours sur le plan écologique, ce système permettrait d'automatiser la fourniture de la vignette Crit'air dans les villes qui l'utilisent. Ce serait également un moyen de sensibiliser les usagers sur la nécessité d'anticiper leur contrôle technique ou de mettre en place des systèmes d'alertes ciblées en cas de circulation alternée.

que les difficultés rencontrées par l'ANTS pour la délivrance des certificats d'immatriculation soient liées à la problématique de la dématérialisation du mode de paiement des taxes. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même si j'ai compris que le ralliement de M. Bocquet à l'amendement de la commission rendait ma tâche particulièrement périlleuse.

Avançons certes vers la numérisation, mais veillons à ce que le poids de la médiation, qui sera certainement nécessaire pour une partie des habitants, ne pèse pas que sur les collectivités territoriales

ce peut être sympathique- on résorbe d'une certaine façon des problèmes d'emploi -, mais, dans des communes relativement éloignées, cette situation est extrêmement préjudiciable pour les personnes qui subissent la fracture numérique. Je mets aux voix

kilomètre. Cet amendement tend à appliquer au superéthanol les mêmes avantages fiscaux que pour l'utilisation du GPL et du GNV, les trois carburants étant alternatifs et bénéficiant d'une fiscalité très réduite par rapport à l'essence ou au gazole. Le fort contenu en bioéthanol du E85 le différencie des deux autres carburants à eux, fossiles. L'abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du superéthanol E85 répond au caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol. Le carbone biogénique est effectivement renouvelable en un an, alors que le carbone fossile l'est dans un délai extrêmement long. Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol. Le bioéthanol réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66 % en moyenne en Europe. de loi de finances rectificative pour 2016 pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié et entrera en vigueur au 1 janvier 2018. Or, pour l'heure, l'exonération de douze trimestres de la TVS est ouverte aux seuls véhicules hybrides électriques-superéthanol. Cette disposition est parfaitement subjective et contraire aux engagements pris en matière de réduction de CO2 et de particules, dans le cadre de la COP21 et, aujourd'hui, de la COP23. Cet amendement a donc pour objet de combiner le superéthanol également au GNV ou au GPL. Le coût de cette exonération pour le budget pour 2018 serait faible par rapport au bénéfice attendu.

d'accession sociale à la propriété situées dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain, le taux réduit de TVA à 5,5 % pourrait s'appliquer dès la signature du protocole de préfiguration à la convention.

ou d'impôt sur les sociétés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE. Cette clause, qui était de un habitant de ZFU pour cinq employés de 1997 à 2002, est passée de employés en 2002. En 2011, le Gouvernement a fait passer cette clause d'embauche locale à un pour deux salariés. Ce durcissement de la clause d'embauche à 50 % a engendré de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs, ce qui a fait sortir nombre d'entreprises du bénéfice de ce dispositif. C'est pourquoi cet amendement vise à revenir à une clause d'embauche locale de un pour trois salariés.

Cet amendement prévoit que la construction d'immobilier d'entreprise et le recyclage de friches en immobilier d'entreprise bénéficient, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires entrepreneurs élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L'objectif est de favoriser la production d'immobilier d'entreprise dans ces quartiers.

L'article 28 prévoit le report d'un an de la date d'entrée en vigueur dans les départements d'outre-mer du monopole de la vente de tabac au détail aux commerçants titulaires d'une licence accordée au nom du conseil départemental.

! -, le Gouvernement est convaincu que les départements d'outre-mer ont besoin d'un délai supplémentaire d'un an pour mettre en place une politique pluridimensionnelle en matière d'encadrement de la vente en détail du tabac. Ce report répond sinon à une urgence, en tout cas à une approche particulière et adaptée aux enjeux sociaux de ces territoires, qui doivent être promus.

Il convient de prendre en considération les conséquences extrêmement négatives du maintien du taux de TVA à 10 % sur le développement des parcs zoologiques, l'emploi, voire la survie de certains parcs.

Beauval est pourtant classé parmi les dix plus beaux zoos du monde. En outre, je tiens à rappeler les missions d'intérêt public des parcs zoologiques définies dans l'arrêté du 25 mars 2004, au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l'éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l'activité de recherche scientifique. La naissance médiatisée du bébé panda Yuan Meng à Beauval cet été prouve le rôle fondamental des zoos dans la protection des espèces menacées. Ce nom, Yuan Meng, signifie la réalisation d'un rêve ou d'un souhait. Mes chers collègues, il vous est donc proposé de revenir à ce souhait : un taux de TVA à 5,5 % pour les parcs zoologiques. Pour

L'article 29 fusionne plusieurs procédures de recouvrement forcé, aujourd'hui très nombreuses,

qui ne sont pas repris dans la nouvelle version de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Autant la commission est favorable sur le fond à l'unification des procédures, autant elle souhaite conserver une obligation de notification.

Une difficulté se pose. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales définit le champ des contestations relatives au recouvrement des créances publiques. À ce titre sont visées les contestations relatives à l'obligation « au » paiement, qui est le terme juridiquement adéquat. Viser des contestations relatives à l'obligation « du » paiement nous paraît impropre juridiquement, la jurisprudence retenant le terme de l'obligation au paiement ou de l'existence de l'obligation de payer.

nous sommes favorables à l'unification, autant nous ne pouvons souscrire à la restriction du champ des recours des contribuables. C'est l'objet de cet amendement. Gouvernement ? Pour le Gouvernement, la mention « sur l'obligation au paiement » est suffisamment large pour inclure toutes les contestations autres que celles qui remettent en cause le calcul et l'assiette de l'impôt, qui sont les seules exclues expressément par la rédaction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable

Gouvernement ? Cet encadrement est lié à la création de la saisie administrative à tiers détenteur, qui entre en vigueur à compter du 1 janvier 2019. C'est la raison pour laquelle, souhaitant un alignement de dates, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement se fixe deux objectifs avec l'abaissement du plafond au-dessus duquel il serait interdit de payer en numéraire. Le premier est un objectif de simplification et de dématérialisation. L'abaissement du plafond en 2014 montre que cela porte ses fruits. Le second objectif tient aussi à la sécurité des régisseurs,

du plafond au-dessus duquel il sera interdit de régler en numéraire. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement renvoie à un tel décret. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Je veux juste souligner que, si les dispositions prévues par le Gouvernement étaient adoptées, un pas supplémentaire serait franchi vers le rêve ultime de l'administration qui est de faire disparaître les règlements en numéraire pour nous contrôler encore un peu plus dans notre vie quotidienne.

de réduire les délais de paiement : en France, on estime à plus de 600 milliards d'euros le crédit interentreprises, c'est-à-dire les dettes réciproques entre les entreprises provoquées par les délais de paiement. La réduction des délais de paiement répond à la première préoccupation des créateurs d'activité, en particulier les PME et les TPE : l'amélioration de la trésorerie est un véritable indicateur de la santé économique d'une entreprise. Par ailleurs, l'amélioration des délais et la traçabilité de la facturation permettent d'améliorer la qualité de la relation entre les entreprises et leurs clients : les problèmes liés à la facturation sont l'un des principaux motifs de saisine du médiateur des entreprises. Le portail de facturation électronique Chorus Pro a été créé par l'État, plus exactement par l'Agence pour l'informatique financière de l'État, l'AIFE pour permettre à la sphère publique- État, collectivités territoriales, établissements publics -de contribuer à l'amélioration de ses propres délais de paiement au bénéfice de ses fournisseurs. Cette solution mutualisée a connu ses premières étapes de déploiement avec succès, et sa généralisation À titre d'exemple, 99 % des collectivités locales ont reçu et téléchargé une facture au moyen de la solution Chorus Pro. En 2017, plus de 10 millions de factures transiteront par ce biais, et environ 100 millions à terme. Toutes les grandes entreprises ont aujourd'hui l'obligation d'adresser leurs factures aux entités publiques Chorus Pro ; cette obligation s'appliquera également aux ETI dès janvier 2018, aux PME et aux TPE d'ici à 2020. On peut noter, alors qu'on s'interroge sur la meilleure manière de moderniser nos administrations, qu'il s'agit d'un projet à fort impact ayant respecté des délais pourtant courts : l'obligation d'utiliser Chorus Pro a été adoptée dans cet hémicycle en 2014 et son entrée en vigueur est intervenue en 2017, obligeant la solution à être conçue et déployée en moins de trois ans. L'État doit toutefois se montrer exemplaire, et c'est le sens du présent amendement : la DGFiP adresse aujourd'hui 30 000 titres de perception aux collectivités locales au moyen d'un envoi physique en utilisant les services postaux, car la loi ne lui permet pas d'utiliser Chorus Pro dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes. Veuillez conclure,

de prévoir le séquençage des faits générateurs entre le conventionnement, les études d'impact, l'évaluation archéologique et le diagnostic. Il est question d'ajouter au titre des exemptions de paiement

Nous partageons tous l'objectif de préservation de notre patrimoine archéologique et le Gouvernement est évidemment attaché à ne pas négliger le patrimoine maritime, y compris dans nos ports. Les amendements que vous proposez visent à créer des régimes d'exception ou d'exonération.

comme l'agriculture et fait donc l'objet d'une exonération. Je sais que c'est un sujet de préoccupation ; il est par conséquent utile de le clarifier. Nous considérons qu'en créant de tels régimes d'exception ou d'exonération, ces amendements risquent en revanche d'affaiblir la protection du patrimoine, dans la mesure où ils portent atteinte au principe selon lequel

Rapin. Cet amendement vise à fixer le moment auquel doit être réalisée l'évaluation archéologique. Il est proposé de mettre en oeuvre un protocole d'évitement des biens culturels maritimes qui pourra être intégré à l'étude d'impact.

des travaux, à des éléments du patrimoine archéologique. La définition d'un protocole d'évitement nécessite impérativement d'avoir préalablement détecté, identifié et caractérisé ces éléments du patrimoine archéologique présents sur l'emprise du projet. C'est précisément l'objet de l'évaluation archéologique. Le protocole d'évitement

Monsieur le rapporteur

du Gouvernement ? Le droit en vigueur permet déjà un fractionnement lorsque les travaux sont réalisés par tranches et que celles-ci sont prévues dans l'autorisation administrative. La rédaction de cet amendement nous semble trop large pour être opérante. Cependant, nous examinerons les possibilités techniques qui permettraient d'annualiser la perception de la RAP pour certaines catégories de travaux. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra

calcule les attributions de compensation. Certaines compétences des EPCI ont pu initialement être évaluées par des CLETC selon des méthodes et des règles de majorité qualifiée des conseils municipaux

l'adoption de l'amendement que vous proposez nous paraîtrait de nature à complexifier le système de calcul de l'attribution de compensation et celui de l'évaluation du montant des charges transférées, ce qui n'est évidemment pas votre objectif. Par ailleurs, vous l'avez dit, monsieur le sénateur Raynal, est partiellement satisfait par la possibilité de fixer librement le montant de l'attribution de compensation, dont les modalités ont été simplifiées par la loi de finances initiale pour 2017. Je me

principe, tout vote positif au sein du conseil. C'est la raison pour laquelle nous avons transformé le vote à l'unanimité du conseil communautaire en un vote à la majorité qualifiée, mais en assortissant cette modification

La séance est reprise.

que, pour être applicables l'année suivante, les délibérations prises par les EPCI ou les communes affectataires de la taxe doivent être prises avant le 1 octobre, date limite de droit commun en matière de fiscalité directe locale.

Ce département est confronté à nombre de défis et la suppression de l'APL-accession briserait la dynamique locale en faveur de l'accession sociale à la propriété.

cette aide est absolument indispensable pour multiplier les dispositifs de construction de logements et leur donner un coup de pouce salvateur. Mayotte doit faire face à une demande de construction particulièrement importante, qui ne fera que croître dans les années à venir. À la différence du du reste du territoire national, la collectivité connaît, en effet, une démographie galopante. Pour rappel, l'accroissement naturel mahorais est estimé à 3,1 par an, quand la moyenne française est de 0,4 %. Autre signe du besoin à venir en logements : plus de 46 % de la population de l'île a moins de 15 ans,

en énergie. Lorsque les critères sont remplis, les taux réduits s'appliquent à l'ensemble des consommations du site ou de l'entreprise. Certaines entreprises, qui n'exercent pas elles-mêmes d'activité industrielle proprement dite, peuvent entrer mécaniquement dans le champ d'application des taux réduits, au seul motif qu'elles exploitent des installations secondaires dont l'activité est susceptible de relever des sections B et E de la nomenclature d'activités et de produits français. L'amendement n° 70 avait pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité accordés à raison d'une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d'une installation industrielle caractérisée

de soumettre l'application de cette disposition à un décret. Ce décret permettra, à l'issue d'une concertation avec les acteurs économiques concernés- producteurs d'électricité, Conseil supérieur de l'énergie ... -de garantir que les effets de bord qui étaient craints par certains,

pas d'opposition de principe sur l'idée de modifier le code des douanes et son article 266 L'amendement apporte des réponses de ce point de vue, puisqu'il prévoit le renvoi à un décret

Nous n'avons pas eu le temps de mener la discussion interministérielle, monsieur le président ... Plus sérieusement, j'ai oublié, et j'aurais dû commencer par là, de vous demander de bien vouloir excuser le Gouvernement pour ce dépôt d'amendement extrêmement tardif dans la discussion. Vous avez compris qu'il y avait eu un certain nombre de discussions dans la journée qui expliquaient cela. Je remercie M.

de l'ordre de 50 %, du fait de la multiplication des allocataires et de l'augmentation de 10 % au-delà de la revalorisation basée sur l'indice des prix à la consommation

que les fonds de 2016 versés au titre du RSA en 2017 soient pris en compte dans le calcul pour le fonds de soutien de 2017, puisque le fonds de soutien de 2016 lui-même a été voté en 2017. Je ne sais pas si je suis très clair, mais, en tout cas, les comptables s'y retrouveront ! Je suis

ces difficultés, qui peuvent poser des problèmes de coordination ou d'imprévisibilité des ressources dont bénéficient les départements. Comme vous l'avez dit, l'attribution d'un fonds de secours en fin d'année ne peut pas véritablement être anticipée et intégrée lorsque les départements ont à rendre des arbitrages budgétaires. Vous le savez, la Conférence nationale des territoires s'est tenue hier. Parmi les dispositions examinées, il y a la contractualisation entre l'État et les collectivités pour modérer le rythme d'évolution de la dépense publique, particulièrement de la dépense des collectivités locales. L'objectif du Gouvernement est que l'évolution des dépenses des départements soit limitée à 1,2 % par an pendant les trois ans qui viennent. En revanche, et cela fait écho à vos préoccupations en matière de financement des allocations individuelles de solidarité, les AIS, il a été d'ores et déjà indiqué par le Premier ministre- le Gouvernement a d'ailleurs déposé des amendements sur ce point dans le cadre du débat qui se tient actuellement à l'Assemblée nationale que, parmi les critères d'évaluation et pour la définition du périmètre des dépenses concernées par la limitation à 1,2 % seraient neutralisées les dépenses

dans les critères de répartition de cette enveloppe exceptionnelle. Au-delà des AIS, on sait que la prise en charge des mineurs non accompagnés est un vrai problème pour les départements. Surtout, elle est extrêmement variable d'un département à l'autre, notamment en fonction de leur situation géographique. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale souhaitait que le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par les départements figure aussi au rang des critères de répartition de cette enveloppe de 100 millions d'euros. L'amendement vise simplement

que seront imputées dans les dépenses vérifiées, ou en tout cas tenues à une maîtrise de leur augmentation à 1,2 %, uniquement celles qui correspondent à l'augmentation entre 0 % et 2 % ; l'augmentation de 2 %

avons bien examiné la part de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, la TICPE, qui était dévolue aux régions et aux départements pour couvrir une partie des transferts de compétences et de charges que les lois de décentralisation ont pu opérer. Très sincèrement,

des mineurs étrangers isolés- je ne peux pas les appeler mineurs non accompagnés, tellement ils sont bien accompagnés jusqu'à nos services sociaux par les filières qui s'engraissent sur le dos de nos contribuables ! -, les départements aujourd'hui n'en peuvent plus. Je dois dire enfin que le montant de 100 millions

d'aboutissement intéressant pour les départements. La situation devient dramatique et il faut vraiment que le Gouvernement se dépêche de parler sérieusement avec les départements ! La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

à partir du moment où certaines compétences qui sont transférées étaient exercées soit par un syndicat fiscalisé, soit par un syndicat non fiscalisé. Il en résulte une inégalité. Cet amendement a donc

en leur permettant de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. L'article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion

On sait que cela se fera plutôt la semaine prochaine, une fois encaissée la contribution exceptionnelle des grandes entreprises prévue par le collectif de novembre : une petite affaire de 5 milliards d'euros, sans correctif possible, qui frappe des entités économiques pesant 1 620 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

que bien des attentes et des besoins demeurent sans couverture. La retenue à la source a constitué une des clefs de ce débat. Notre groupe demeure clairement opposé à cette réforme totalement inutile à notre pays du point de vue des rentrées fiscales.

vote. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous venons de finir l'examen de ce collectif budgétaire de fin d'année.

Comme chaque année, les délais très contraints ont rendu difficile un examen approfondi et éclairé de dispositions qui sont à la fois très diverses et Si des mesures bienvenues, comme la généralisation de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes, l'interdiction des réservations en ligne par cartes prépayées, ou encore la réduction des intérêts moratoires, ont été conservées, la Haute Assemblée est revenue sur l'une des principales réformes contenues dans ce texte, à savoir le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Nous regrettons également certains aménagements fiscaux, notamment à l'impôt sur la fortune immobilière, et d'autres modifications du texte préférées aux amendements déposés par notre groupe. Comme

pour explication de vote. Ce projet de loi de finances rectificative n'échappe pas à la tradition : il compte maintes mesures techniques qui seront utiles à de nombreux secteurs professionnels. Je voudrais souligner l'adoption de plusieurs propositions émanant de la commission des finances en matière de fiscalité

que, sur de nombreux sujets, nous attendons de vrais engagements, une action volontariste en matière de réduction de la dépense publique, et des réformes structurelles qui seules permettront de réduire durablement notre déficit

Le scrutin est ouvert.